La séance est reprise. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, aujourd'hui, a été rendu à Nîmes un hommage aux trois secouristes décédés en début de semaine dans l'accident d'un hélicoptère de la sécurité civile dans les Bouches-du-Rhône. Deux d'entre eux servaient au sein de la sécurité civile et le troisième au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Ils ont perdu la vie en portant secours à nos concitoyens frappés par les violentes intempéries qui ont touché le sud-est de la France ces jours derniers. En votre nom, je souhaite associer notre assemblée à cet hommage, saluer leur mémoire et leur engagement, comme celui de tous les personnels des services de secours, et assurer leurs familles de nos condoléances les plus attristées. Nous poursuivons l'examen,

Cet amendement tend à remédier à l'iniquité et aux aberrations du régime fiscal relatif à la prise de garanties immobilières dans le cadre des mesures conservatoires. La superposition de taxes et contributions diverses que doivent acquitter les créanciers qui veulent prendre une mesure conservatoire sur les biens immobiliers de leurs débiteurs est dépourvue de toute légitimité et constitue un frein à l'obtention d'une telle mesure. Depuis un édit de Louis XV du 17 juin 1771, et jusqu'au 1 janvier 2013, existait ce qu'on appelait un conservateur des hypothèques. Cette « fonction » a été supprimée par l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques. Il est dès lors choquant que la suppression des conservateurs des hypothèques n'ait pas eu d'incidence directe sur le coût des hypothèques conservatoires.

l'impôt sur la fortune immobilière, et en le remplaçant par l'IFI, l'impôt sur la fortune improductive, pour le coup, le ruissellement sera sans doute réel. En effet, si l'on taxe les liquidités

Depuis le remplacement de l'ISF par l'IFI, le portage foncier n'est plus attractif pour les investisseurs, dans la mesure où l'impôt sur la fortune immobilière marginalise le foncier

d'appartenir à la même société, d'épargner pour eux ou pour leurs enfants, de constituer un patrimoine familial et personnel, ce qui était autrefois la base de la transmission dans ce pays. Ne cassez donc pas les bases, parce que vous ne parviendrez pas à en créer de nouvelles.

notre part, nous avons réduit la base taxable de l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que nous estimions qu'une partie de ce qui était taxé- comme l'ont démontré assez largement des économistes de différents bords

ou d'enseignement artistique, publics et privés, des organismes d'insertion et d'aide à la création ou à la reprise d'entreprises en difficulté, des fondations universitaires, de l'Agence nationale de la recherche, etc.

À cet égard, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un cadre favorable au développement de la filière bois, fondé sur des objectifs très volontaires pour mobiliser la ressource d'ici à 2035. Aussi, cet amendement vise à pérenniser l'un des leviers encourageant l'investissement forestier, le DEFI forêt. C'est un outil que nous avons déjà reconduit en loi de finances, mais le pérenniser permettrait de donner davantage de visibilité aux acteurs de la forêt. fiscal permet de concourir à la lutte contre le morcellement de la propriété forestière, au développement des travaux forestiers, ainsi qu'à l'organisation économique du secteur. Il serait également souhaitable de l'aménager fiscalement

car il permet de procéder à des remembrements forestiers sur l'ensemble de nos territoires forestiers, que nous savons très morcelés. J'ajoute qu'il oblige à mettre en place un document de gestion durable, ce à quoi, on le sait, nos concitoyens sont très attentifs.

rectifié vise à étendre l'avantage fiscal aux agrandissements des propriétés forestières les plus vastes, par l'acquisition de petites parcelles, ce qui n'est pas l'objectif du dispositif.

Cet amendement de Joël Labbé vise à créer une taxe d'un montant de 1,5 % sur les dépenses publicitaires des produits alimentaires. Elle serait destinée au financement de la transition écologique de l'agriculture.

entre la commune d'implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d'implantation. Cela permettrait une plus juste répartition entre les collectivités locales concernées.

François Bonhomme. Cet amendement a pour objet de permettre aux musées associatifs qui interviennent en matière de conservation des objets du patrimoine rural, paysan et artisanal, ainsi que des arts et des traditions populaires, d'être exonérés de manière permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

d'intérêt général. Les associations propriétaires de musées ne font pas ou font peu de bénéfices. Ce sont donc autant de moyens financiers qui ne peuvent pas être investis dans la sauvegarde du patrimoine local ou dans le déploiement de nouvelles formes d'accessibilité à la culture.

ayant acquis ou louant les locaux dans lesquels ils assurent des activités de soins de premier recours et, le cas échéant, de deuxième recours. Il s'agit ainsi de mettre fin à une rupture d'égalité entre deux types de structures ayant le même objet. Les professionnels libéraux exerçant dans des structures mises en place par les collectivités locales bénéficient de conditions d'exercice et de loyer bien plus avantageuses que les professionnels de santé exerçant dans des structures privées. Pourtant, ces derniers sont soumis aux mêmes obligations d'accès aux soins et aux mêmes conditions tarifaires.

technologique, contre 1 607 euros par an au 1 janvier 2016. Si un même point haut est équipé d'une antenne 2G, d'une antenne 3G, d'une antenne 4G et, à partir de 2020, d'une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois. Afin de tenir compte des difficultés particulières d'implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l'article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l'IFER. de juin 2017, selon les chiffres de la Fédération française des télécoms, 3 166 nouveaux sites 4G ont été activés en zone de montagne pour atteindre un total de 6 258. L'exemption d'IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne, qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l'altitude et au climat. Afin d'accélérer la généralisation de la 4G en montagne d'ici à la fin de l'année 2022 prévue par le mobile, le présent amendement vise à proroger au 31 décembre

contradictoire. Plus les opérateurs déploient des sites mobiles qui participent à l'amélioration de la couverture numérique du territoire, plus ils implantent des technologies de dernière génération qui augmentent leur charge fiscale. Le produit de l'IFER mobile a ainsi connu une hausse continue qui pèse sur leur capacité d'investissement et freine les déploiements. L'arrivée de la 5G risque d'amplifier très fortement le phénomène et d'inciter les opérateurs à étaler les déploiements dans le temps, sous peine de faire exploser la facture fiscale.

Chaque opérateur devra ainsi déployer au minimum 12 000 sites 5G d'ici à 2025, soit un total de 48 000 sites. Sans l'introduction d'une modération fiscale spécifique à la 5G, l'IFER mobile augmentera mécaniquement de 80 millions d'euros en 2025

et sa généralisation rapide sur l'ensemble du territoire. Aussi, le présent amendement vise à introduire une exemption d'IFER mobile pour les stations radioélectriques 5G qui seront construites entre le 1 janvier 2020 et le 31 décembre 2025, afin de garantir les conditions d'un déploiement rapide et effectif.

Enfin, si ce taux de 5,1 % devait paraître confiscatoire, ou inquiéter certains, les amendements suivants

d'État, pas à nous, pas ici ! Comme dirait le président Marseille, ce n'est pas entre romanichels qu'on se raconte la bonne aventure

Par ailleurs, afin de substituer progressivement la taxation des réseaux cuivre à celle des réseaux FTTH, il est prévu de maintenir trois années de plus cette exonération pour les réseaux FTTH labellisés « zones fibrées » au sens de l'article L. 33-11 du code Avec un tel système, l'accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan Très haut débit ne seront pas pénalisées.

dans le secteur privé, 29 % des salariés ont pratiqué le télétravail de façon occasionnelle ou régulière en 2018, contre 25 % l'année précédente, selon une enquête de l'IFOP. La France est en retard,

Par ailleurs, dans le secteur privé, 15,5 % des établissements de plus de dix salariés ont mis en place le télétravail. Pour lutter contre la pollution liée aux allers-retours, mais aussi pour pallier les effets des grèves que nous subissons les pouvoirs publics encouragent les entreprises à avoir recours au télétravail. Le Gouvernement a ainsi assoupli la réglementation encadrant la pratique à l'automne 2017. Une étude récente de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux a montré que le télétravail, en économisant des déplacements, a permis une a permis une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 3 % à 5 %. Cette proposition vise donc à répondre à ces enjeux et à simplifier et à sécuriser le calcul des effectifs concernés par l'exonération du versement mobilité. En effet, ce dispositif est conforme à la règle fixée par l'article

% dans le cas où, sur le territoire concerné, un projet d'infrastructures de transport collectif en mode guidé a obtenu une déclaration d'utilité publique. Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de l'offre de transports collectifs dans les territoires. Il est aujourd'hui indispensable de développer les transports les transports en commun dans les zones urbaines, au-delà de la seule Île-de-France, afin de répondre aux enjeux environnementaux et de mobilité des populations. En effet, le taux du VT a augmenté ces dernières années en Île-de-France, notamment du fait de la loi de finances pour 2018. Cependant, il n'y a pas eu de revalorisation du taux du VT en province. Cet amendement tend donc à corriger cette disparité à donner davantage de flexibilité aux autorités organisatrices de la mobilité, afin d'encourager le développement de l'offre de transports collectifs structurants en province.

des projets acceptés par l'État au travers d'une déclaration d'utilité publique.

Le scrutin est ouvert.

(FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle. Les prélèvements ou les reversements des communes et EPCI au titre du FNGIR sont calculés sur la base d'une comparaison des ressources fiscales avant et après la réforme de 2010. Conformément à l'article 40 de la loi de finances pour 2012, qui précise que, à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement correspondent aux montants perçus ou versés en 2013, les montants des prélèvements ou reversements au titre du FNGIR sont désormais figés, sans perspective de mise à jour. Précisément, toutes les évolutions économiques des territoires postérieures à 2010 ne sont pas prises en compte dans le calcul. Il ne s'agit pas ici de simplement compenser les conséquences fiscales de la fermeture d'une entreprise pour la collectivité territoriale concernée, mais de permettre une révision des bases de calcul de sa contribution au FNGIR en tenant compte de sa nouvelle situation. Cet amendement prévoit qu'un prélèvement

charges sociales et fiscales, bonification de subventions ou dotations, assouplissements réglementaires -arriveront à échéance à la fin de 2020. Les auteurs du rapport proposent une prolongation de ce dispositif avant une refonte prévue pour Parallèlement, nos collègues députés ont mené l'an passé une mission « flash » sur le sujet, qui conclut, comme bien d'autres études, au faible effet incitatif du dispositif actuel sur les territoires concernés, notamment en matière de croissance, d'emploi et de création nette d'entreprises. Les raisons de cette faible efficacité tiennent principalement au saupoudrage des moyens accordés,

et à l'urgence d'agir contre le changement climatique, il est de la responsabilité du législateur de mettre en place tous les outils possibles pour faire évoluer notre modèle productif et, en même temps, lutter contre les effets d'agglomération, qui conduisent à la concentration de l'activité économique dans les métropoles.

Prélevées sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur, les recettes de la taxe affectée à la filière française du cuir proviennent principalement des grandes maisons de luxe et profitent en priorité aux PME et TPE de la filière, des actions d'accompagnement mises en oeuvre par le CTC. Cette taxe n'est pas considérée par les acteurs de la filière comme une taxe de production pesant sur la compétitivité des entreprises, mais au contraire comme un investissement mutualisé au profit de l'ensemble de celles-ci, reconnu et validé par la profession. Fixé jusqu'en 2019 à 0,18 %, son taux n'avait jamais été remis en cause par les acteurs de la filière. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2019, un système de fourchette de taux a été introduit. Désormais, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur de cet intervalle. La définition d'un taux adapté correspondant aux besoins réels du CTC ne peut faire l'économie peut faire l'économie d'une concertation avec les acteurs de la filière. Aussi, dans son rapport intitulé « Plateformes d'accélération vers l'industrie du futur : organisation, missions et financements des centres techniques industriels (CTI) et comités professionnels de développement économique (CPDE) », la députée Anne-Laure Cattelot recommandait de mettre les filières au centre de la décision, en préconisant que les assiettes des taxes affectées soient fixées par arrêté pris sur proposition des organisations professionnelles concernées pour maintenir une bonne correspondance entre cotisants et bénéficiaires des actions collectives. Cet amendement, qui tient particulièrement à coeur à ma collègue Catherine Dumas, prévoit que le taux de la taxe affectée à la filière française du cuir puisse être révisé chaque année, sur proposition des organisations professionnelles, par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Quel est l'avis de la commission ?

de séjour. Contrairement à la taxe de séjour « au réel », les sommes dues par les logeurs au titre de la taxe de séjour forfaitaire doivent être intégrées à la base d'imposition à la TVA depuis 1994. Ainsi, pour 100 euros de taxe de séjour versés à la commune, le régime forfaitaire impose à l'hôtelier

Arnaud Bazin. L'article 162 de la loi de finances pour 2019 avait prévu, pour les communes n'ayant pas délibéré dans les temps, une reconduction automatique des tarifs de la taxe de séjour applicables en 2018 et, surtout, un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés pour les collectivités concernées se retrouvant dans l'impossibilité matérielle de délibérer au titre de l'année 2019. Cet amendement vise à prolonger à titre exceptionnel en 2020 cette faculté de reconduction du tarif par défaut de 1 du coût par personne de la nuitée pour les hébergements non classés, prévue pour les communes n'ayant pas délibéré dans les délais prescrits par la loi. Quel est l'avis

vise simplement à réduire le coût d'utilisation des moyens de paiement dématérialisés- cartes bancaires, virements et applications sur portable -, afin d'en favoriser l'usage, et ce sans seuil minimum d'achat, au moyen d'une compensation fiscale. Quel est l'avis de la commission ?

ou autres emplacements de même nature. Or seuls quelques espaces isolés sur ces hippodromes peuvent être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales, mais en aucun cas

services fiscaux départementaux. Quel est l'avis du Gouvernement ? Il n'y a pas de raison qu'il y ait des discordances d'un endroit à l'autre. En tout cas, cela doit pouvoir être rectifié.

La réforme de la taxe professionnelle a déstabilisé l'indépendance et l'autonomie de gestion des collectivités territoriales, sachant qu'elle représentait 34 % de leurs ressources.

L'imposition économique ne pèse plus que 110 euros en moyenne par habitant en 2017, contre 330 euros pour la Ce déséquilibre résulte d'un ensemble de dégrèvements, exonérations, niches, compensations en faveur des entreprises. Nous proposons donc de modifier la base de la CET afin qu'elle prenne en compte la réalité économique et les choix de construction capitalistique des entreprises, comme la suraccumulation du capital du capital financier. Ajouter à la CET en tant que base imposable les actifs financiers figurant au bilan des entreprises assujetties permettrait, d'une part, d'abonder les ressources des collectivités territoriales, et, d'autre part, de contribuer à modifier les choix de gestion des entreprises en faveur de l'emploi et de l'investissement productif. Quel

à M. Julien Bargeton. Nous le savons, la France se distingue par un niveau élevé d'impôts sur la production, c'est-à-dire sur la propriété, sur l'utilisation des terrains, sur les actifs de production comme les machines ou sur la masse salariale.

C'est surtout beaucoup plus que nos voisins : 0,5 % de la valeur ajoutée en Allemagne, contre 3,6 % en France. Les analyses économiques ne manquent pas pour décrire les distorsions qui sont induites par ces impôts de production, notamment dans la chaîne de production ou sur ce que les économistes appellent la productivité des facteurs.

retrait. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Le présent amendement a pour objet de permettre la modulation de la Tascom dans les communes signataires d'une convention ORT en prévoyant la possibilité, pour la collectivité ou l'EPCI, soit de la réduire à hauteur du montant des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien du local assujetti, soit d'en exonérer totalement les entreprises situées dans le périmètre ORT. Cette exonération pourrait être conditionnée à la remise en état du local pour contribuer à l'embellissement des centres-villes. À l'inverse, la collectivité ou l'EPCI pourrait décider son augmentation de 30 % en dehors du périmètre ORT pour les commerces d'une surface de vente supérieure à 2 000

Monsieur Bonhomme, Même si, formellement, cette déductibilité n'est pas entièrement supprimée, puisque l'article qui la prévoit, à savoir l'article 200 du CGI, est toujours en vigueur, le dernier paragraphe la prive désormais d'effet et la rend caduque,

si les champs d'application de ces deux taxes sont très proches, elles diffèrent quant aux exonérations applicables. S'agissant de la taxe sur les bureaux, votre demande est en grande partie déjà satisfaite, dans la mesure où les salles de soins ou d'examen des maisons médicales en sont exonérées ; ce n'est en revanche pas le cas pour ce qui est de la taxe pour création de bureaux.

et qu'elle permet un effet d'aubaine pour certaines collectivités territoriales. Il faudra, dans le cadre de la remise à plat des modes de financement des collectivités, s'intéresser à cette surtaxe.

La loi de finances pour 2013 a déjà renforcé la taxe sur les logements vacants en augmentant ses taux. Son poids est devenu suffisant pour sensibiliser les propriétaires de logements vacants situés en zones tendues à l'incidence socioéconomique de la rétention de logements.

la taxe sur les logements vacants est destinée à financer la politique du logement, l'Agence nationale de l'habitat. Il serait donc totalement injustifié d'en affecter une partie du produit aux communes, sauf à vouloir remettre en cause la politique du logement ; je ne pense pas que telle soit l'intention de la Haute Assemblée. Une telle mesure profiterait non pas à toutes les communes, mais avant tout à celles qui pratiquent des taux élevés de taxe

cet amendement pourrait, à l'inverse, être défavorable aux bailleurs et les conduire à ne pas investir sur le territoire de certaines communes marquées par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. l'on donnait aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale la liberté de délibérer pour mettre en oeuvre une exonération totale de TFPB, le maintien d'une compensation par l'État ne se justifierait plus. Cette mesure serait en outre sans effet sur les exonérations déjà accordées pour la durée restant à couvrir. L'avis du

(ANRU), la nouvelle construction ne peut plus, depuis 2017, bénéficier des régimes d'exonération de taxe foncière prévus pour ces opérations si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux.

Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, demeurent soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Or l'administration fiscale assimile parfois ces locaux à des établissements industriels et applique par conséquent l'imposition sur la valeur brute des bâtiments, et non sur l'importance de l'activité qui y est exercée. Cette situation est pénalisante pour des bâtiments abritant des activités qui ne s'exercent que de manière saisonnière ou ponctuelle. C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement, qui vise à étendre à ces locaux les dispositions applicables aux locaux servant à l'hébergement des salariés saisonniers

Il est ici question de la situation d'un acquéreur qui donne à bail à construction un terrain à bâtir. Nous souhaitons sécuriser les projets immobiliers et éviter une double taxation

? L'amendement est déjà satisfait en l'état du droit. En effet, le tarif de 125 euros en sus de la TVA reste acquis dès lors que les travaux de construction sont réalisés dans un délai de quatre ans, que ce soit par l'acquéreur-bailleur ou par le preneur.

pour les immeubles neufs situés en zones tendues A et A . Autant le dispositif existant se justifie pour dynamiser la construction de logements, autant il est tout à fait inutile

Afin de favoriser les opérations d'accession à la propriété destinées aux ménages modestes, le présent amendement vise à permettre aux conseils départementaux qui le souhaiteront d'exonérer de droits d'enregistrement les ventes de logements réalisées dans ce cadre, sous réserve du respect des conditions qui s'imposent aux organismes d'HLM en matière d'accession sociale à la propriété, qu'il s'agisse des plafonds de ressources des accédants, du plafonnement des prix de vente ou encore des garanties de rachat et de relogement. Cette mesure vient compléter l'article 1594 G du code général des impôts, qui prévoit une exonération facultative de droits d'enregistrement pour les ventes de logements locatifs sociaux aux locataires.

Pour soutenir ce dispositif, notre amendement vise à instaurer une exonération facultative, soumise à décision des conseils départementaux, pour les acquisitions de logements réalisées dans ce cadre.

L'accès au logement des personnes en difficulté est une préoccupation majeure du Gouvernement, qui ne voit pas d'obstacle au principe d'une exonération facultative permettant de favoriser des solutions alternatives à l'hébergement d'urgence, comme le recours à l'intermédiation locative des agences agréées. En revanche,il n'est pas envisageable que l'État compense de plein droit les nouvelles exonérations.

Il contribue à limiter les feux de forêt, par la consommation de phytomasses combustibles, ainsi qu'à conserver des milieux naturels de grande valeur, tels que les parcs nationaux, les sites Natura 2000 et les réserves naturelles. À ce titre, c'est une activité reconnue d'intérêt général par l'article L. du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'agriculture de montagne. Toutefois, l'activité pastorale doit faire face à un certain nombre de contraintes liées à la difficulté du terrain et à la présence du loup, espèce dont espèce dont on sait qu'elle est douée de facultés d'adaptation importantes. Le gardiennage permanent est donc un moyen nécessaire de protection des troupeaux, ce qui implique souvent l'embauche de bergers salariés. En montagne, ces bergers sont logés dans des cabanes pastorales ou chalets d'alpage, selon le massif.

sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? La taxe d'aménagement a pour objet d'assurer le financement des équipements publics nécessaires à l'urbanisation. Toute exonération de plein droit porte préjudice aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.

au travers de l'imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER), perçue chaque année. Il n'est donc pas souhaitable de taxer davantage cette forme d'énergie renouvelable. Là encore, on est dans une contradiction : on dit qu'il faut baisser les taxes,

d'exonération ou d'abattement que les constructions nouvelles. La transformation d'un bâtiment agricole en habitation ou en local d'activité peut avoir un impact, en matière d'urbanisme, équivalent à celui d'une construction nouvelle, et ainsi nécessiter un équipement public- renforcement des réseaux ou voirie.

L'artificialisation des terres entraîne la perte d'espaces naturels agricoles et forestiers, mais également la disparition des fonctions biologiques du sol, la perte de services écosystémiques et un étalement urbain générateur d'externalités négatives. La France s'est engagée, le plan Biodiversité du Gouvernement, à atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette. La fiscalité représente un des moyens pour atteindre cet objectif. Néanmoins, certains outils fiscaux vont, encore aujourd'hui, à l'encontre de cette ambition. Pour rendre cohérente la fiscalité avec la lutte contre l'artificialisation, cet amendement prévoit la suppression de l'abattement de 50 % de la taxe d'aménagement pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. Cette mesure est préconisée par le rapport de Guillaume Sainteny sur les aides publiques dommageables à la biodiversité. L'amendement

en dépit d'une demande soutenue et de conditions d'accès au logement particulièrement difficiles dans l'ensemble des zones tendues. La loi de finances rectificative pour 2017 a introduit un dispositif d'abattement exceptionnel sur les plus-values cessions immobilières pour les seules zones A et A . L'exclusion de la zone B1, dont relèvent certaines métropoles régionales, ne se justifie pas, dans la mesure où les besoins de construction y sont également très forts.

2019. À la suite de la dissolution de la chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA), décidée par l'article 26 de la loi de finances pour 2019, et en vue de préserver le régime fiscal en faveur des entreprises de batellerie artisanale immatriculées antérieurement au registre de la CNBA, l'article 48 a pour objet de rétablir, à compter de 2020, le bénéfice de la réduction de base d'imposition de la cotisation foncière pour les entreprises de la batellerie artisanale immatriculées au répertoire des métiers qui disposent de biens passibles d'une taxe foncière et emploient trois salariés au plus. Dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement, l'article 26 de la loi de finances initiale pour 2019 avait supprimé la taxe sur les entreprises de la batellerie artisanale à compter du 1 juillet 2019.

qui perçoivent cet impôt. Cette disposition est contestable pour deux raisons. D'abord, la filière de l'électricité photovoltaïque se développe aujourd'hui à un rythme correspondant à la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l'énergie, en particulier en raison des dispositifs de soutien mis en place par l'État. les collectivités contribuent significativement au développement de l'électricité solaire, en adoptant des règles d'urbanisme favorables au photovoltaïque ou en mettant à disposition du foncier ou des toitures de bâtiments publics. De manière plus générale, elles jouent également un rôle stratégique pour la transition énergétique au travers del'adoption et de la mise en oeuvre des plans Climat et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Le fait de pouvoir bénéficier d'une recette fiscale l'IFER contribue à inciter les collectivités à favoriser le développement de l'électricité photovoltaïque sur leur territoire. En privant celles-ci de plus de la moitié de ces recettes, la mesure pourrait donc avoir un effet contre-productif.

La mesure de baisse de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux photovoltaïques prévue par l'article 48 apparaît souhaitable pour tenir les engagements de la France en matière de développement des énergies renouvelables. Il s'agit d'une mesure équilibrée, qui préserve les ressources des collectivités, puisqu'elle ne s'appliquera qu'aux centrales photovoltaïques mises en service à compte de 2021. En favorisant

pompage (STEP) hydraulique, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, permettent de stocker de l'énergie en pompant l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l'électricité sur le réseau en turbinant l'eau du bassin supérieur lorsque la demande électrique augmente. Aujourd'hui, elles constituent les moyens les plus importants et les plus performants en termes de stockage d'énergie termes de stockage d'énergie d'origine renouvelable. L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux repose sur les moyens de production électrique et est calculée en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP, qui sont, par nature, puissantes, alors même qu'elles ont vocation non pas à produire de l'énergie, mais à constituer une assurance pour le système électrique. Le passage progressif aux énergies renouvelables requiert de relever un défi de taille : celui du stockage durable et massif de l'électricité. Exonérer

de transfert d'électricité par pompage constituent des centrales hydroélectriques à part entière. L'IFER n'est pas le principal frein au développement de cet outil de la transition énergétique. C'est la raison pour laquelle, afin de soutenir les installations permettant le stockage de l'énergie, en vue de sa restitution ultérieure au réseau, le Gouvernement a choisi d'agir sur le tarif tarif d'utilisation du réseau. À ce titre, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte porte à 50 % le plafond d'exonération du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Par conséquent, les amendements me paraissent satisfaits

Elle doit permettre de donner un signal-prix pour des comportements considérés comme polluants et de dégager des recettes permettant de développer des alternatives. Cet outil s'est développé ces dernières années, notamment avec la mise en place de la taxe carbone,

De la même manière, la gestion de l'eau s'est organisée selon un modèle de fiscalité écologique intégralement affectée, les redevances. Ce modèle a été remis en question, en particulier par le plafonnement du budget des agences de l'eau. Le mouvement des « gilets jaunes », qui s'est constitué en réaction à la hausse initialement prévue de la taxe carbone, a toutefois marqué un coup d'arrêt au développement de cet outil. Constatant le manque de transparence dans l'utilisation des recettes de la fiscalité écologique, le manque de dispositifs incitatifs et le manque de dispositifs de protection des Français les plus précaires, une partie de nos compatriotes a massivement rejeté cette fiscalité,

Le Gouvernement partage l'ambition de donner visibilité et stabilité à la fiscalité écologique. Pour cette raison, il s'est engagé dans une démarche de budgétisation verte, dont les objectifs recoupent largement ceux des auteurs des amendements en termes d'utilisation des recettes et de clarification du périmètre de cette fiscalité.

En effet, les évolutions variétales, issues des demandes des consommateurs, nécessitent de pouvoir serrer et conditionner les récoltes dans des bâtiments qui permettent leur saine conservation, afin de préserver leur valeur marchande. Ainsi, les pommes de terre ne peuvent désormais être stockées pendant l'année nécessaire à leur commercialisation

l'administration fiscale remet en cause cette exonération dès lors que l'exploitant agricole réalise des prestations de nature commerciale à titre accessoire. L'administration se fonde sur la jurisprudence du Conseil d'État, qui est venue préciser que cette exonération était réservée à un usage exclusivement agricole. Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au énonce que le développement d'activités accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération de la taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiment spécialement aménagés

est l'avis du Gouvernement ? Le maintien de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments ruraux en cas d'activités accessoires à des activités agricoles est déjà prévu par l'article 129 de la loi de finances pour 2019.

Dans l'attente de la mise en place de nos propositions et de la nouvelle géographie prioritaire voulue par le Premier ministre à travers l'agenda rural, il est impératif de proroger le dispositif actuel Y mettre fin sans avoir mis en place des mesures alternatives en faveur de la ruralité aurait des conséquences graves dans ces territoires. Le présent amendement vise donc à proroger

à donner de la visibilité aux élus et aux acteurs des territoires ruraux, mais aussi pour laisser le temps de travailler sérieusement et sereinement à la mise en place des nouvelles mesures que nous envisageons. Madame la secrétaire d'État,

Mes chers collègues, je m'adresse à vous : si nous adoptions de manière unanime cet amendement pour sauver les ZRR, le vote du Sénat résonnerait dans les territoires ruraux de France comme un message positif et encourageant pour tous les élus qui se battent au quotidien pour préparer la ruralité de demain ! La parole

au nom du sénateur Alain Bertrand, qui avait remis un rapport sur l'hyper-ruralité. Quel

tout en conservant ses intensités de recherche sectorielles, l'effort de recherche des entreprises y serait de 2,7 %, contre 1,4 % actuellement

forme de CIR. Le Gouvernement allemand a compris quelles étaient les difficultés du système français et s'en est inspiré pour concevoir un dispositif tout autre,

de choisir entre l'application de la directive d'harmonisation des législations sur l'impôt sur les sociétés, qui va dans le bon sens en ce qu'elle permet de lutter contre l'évasion fiscale,

pour les très petites entreprises. La très forte augmentation des aides reçues, notamment depuis 2008, n'a eu pour conséquence aucune augmentation de l'emploi scientifique dans ces entreprises. Selon une autre étude tout à fait passionnante réalisée par l'Edhec, la forte

de la Chine et de tous les autres pays du monde. Je ne pense pas, mon cher collègue, que vous puissiez prétendre que la recherche publique suffise à affronter la concurrence

la sagesse des députés, en indiquant que les données demandées sont très difficiles à constituer par les entreprises, ce qui peut aller à l'encontre d'un objectif de simplification. La nature descriptive des informations demandées les rendra, en tout état de cause, difficiles à exploiter statistiquement. J'avais recommandé une approche par sondage, plus exploitable. C'est en ce sens que le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation produit chaque année une large enquête statistique, qui est disponible, sur la R&D des entreprises. Cela étant, on ne peut refuser à des élus de la République d'avoir une vision complète d'un dispositif

vise à faciliter les partenariats entre recherche publique et recherche privée, grâce à une incitation complémentaire. C'est exactement ce que nous voulons faire : un continuum de recherche, de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche appliquée, avec des circulations beaucoup plus fluides entre chercheurs publics et équipes privées. En effet, cela permet d'avoir une

communiste, je l'assume, mais aussi en tant que chercheur et au nom d'une communauté très large, qui ne comprend plus ce dispositif. S'agissant du lobbying, j'ai reçu, comme vous, des myriades de courriels en faveur du CIR

de quelques entreprises choisies de façon aléatoire et compléter le rapport de notre collègue rapporteur de la commission des finances, de façon à avoir un peu plus d'éléments. Et si cela doit passer par la délégation aux renseignements pour que ce soit encore plus confidentiel, soit ! Il y a là une somme d'argent extrêmement

: La parole est à M. Antoine Lefèvre. Cet amendement de Mme Dominique Estrosi Sassone, que nous avons été un certain nombre à cosigner, a pour objet d'obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d'impôt recherche, dans la limite de la moitié de ce montant. Depuis plusieurs années, les fermetures d'entreprises, non pas en raison de la faillite, mais d'un transfert d'activité dans un autre pays, soit pour des coûts de production, soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés, face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l'impôt sur les sociétés 30 % de leurs investissements en recherche et développement. L'esprit de cet amendement est non pas de restreindre un outil d'attractivité, mais de répondre à une réalité rapportée par la Cour des comptes dans une publication de 2013, que je me permets de citer : « passant de 9 800 à 17 900 entreprises. [ ...] Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 million d'euros à 5,7 millions d'euros, soit un quasi triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances. » Or, sans plafond ni contrôle, il est impossible d'en évaluer les abus. Plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement tend à fixer un cadre d'utilisation large du CIR, sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France. Enfin, si l'article 49 a réduit ce crédit d'impôt, le projet de loi n'a pas établi de procédure de contrôle.